Le CNPE a notamment pour mission de proposer au Gouvernement les orientations nationales de politique de protection de la France, dans le but de construire une stratégie nationale. Il assiste par ailleurs le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernent la protection de l'enfance. Il est constitué de plusieurs collèges représentant les institutions, les collectivités, les sociétés civiles, les associations, les administrations, les associations de professionnels et les organismes de formation.

constituerait pas forcément un gage d'indépendance pour le Conseil. On pourrait imaginer qu'un représentant associatif ou un représentant des conseils départementaux fasse l'unanimité pour présider l'organisme. Je vous propose donc de laisser le décret d'application déterminer les conditions de nomination

requérants vers les bons interlocuteurs.

pour objet de tirer les conséquences de la création de cette base de données, en abrogeant l'article L. 225-7 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que les départements transmettent au ministre chargé de la famille les décisions relatives à l'agrément en vue de l'adoption, et qui n'a donc plus lieu d'être. En résumé, nous créons une base nationale

d'améliorer la connaissance sur les phénomènes de mise en danger des mineurs, et de recenser les bonnes pratiques du secteur, ce qui supposera de suivre les conditions de prise en charge des mineurs protégés. Je vous demanderai donc,

le secrétaire d'État, cet amendement vise à clarifier le rôle et à harmoniser les pratiques du référent de l'aide sociale à l'enfance, afin d'améliorer l'accompagnement des enfants confiés à l'ASE sur l'ensemble

À cet égard, il doit être en mesure de diagnostiquer les insuffisances, et, au vu des besoins identifiés et des réponses apportées, de proposer des ajustements. Les corrections qu'il préconisera doivent permettre d'enrayer l'affaiblissement du dispositif, lorsqu'il se traduit notamment par des réponses par défaut. La

afin d'« organiser les relations entre les acteurs locaux » et de « faciliter la mise en oeuvre de la stratégie nationale et des schémas départementaux de prévention et de protection de l'enfance

Favreau. Cet amendement a pour objet de permettre aux représentants des services départementaux en charge du handicap de siéger dans le comité départemental

Il est essentiel qu'elles le soient, dans la mesure où elles remplissent une mission d'aide aux jeunes admis à l'aide sociale à l'enfance. Leur expérience et leur expertise s'avéreront indispensables pour garantir la pertinence de ces nouveaux comités.

La liste des représentants au sein des comités départementaux pour la protection de l'enfance nous semble effectivement lacunaire, en regard, d'ailleurs, de la composition du Conseil national de la protection de l'enfance, que ce projet de loi institue.

? La présence de ces associations serait pertinente du fait de leur connaissance directe des conditions d'accueil et de leur activité auprès des personnes admises ou ayant été admises dans un service de l'ASE.

C'est le principe même de la démocratie, défini par Rousseau dans le chapitre VI du livre II du par la formule : « Le Peuple soumis aux lois en doit être l'auteur. Il en va ainsi du principe d'autonomie, selon lequel ceux qui subissent la loi et les politiques publiques, ceux qui sont directement concernés par elles doivent être les premiers organisateurs de ces politiques.

Au même titre que les services de l'État, de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'éducation nationale, de l'agence régionale de santé, des organismes débiteurs des prestations familiales, des professionnels de la protection de l'enfance

la caisse d'allocations familiales. Nous proposons également que ce comité comprenne des personnes ayant fait partie du système de protection de l'enfance. Il nous semble effectivement important de recueillir l'avis et les conseils des personnes ayant été placées ou ayant fait l'objet de mesures d'assistance.

partager des informations couvertes par le secret professionnel. Il ne me paraît pas opportun de procéder à cet ajout, même si la consultation et l'association de ces personnes pourraient être très utiles, notamment par le biais des ODPE. L'avis est défavorable sur les deux amendements.

sur la situation de la protection de l'enfance dans le territoire. Ces informations permettront d'améliorer la politique de protection de l'enfance sur l'ensemble du pays, par des analyses pointues, des vérifications qualitatives

La production de données au niveau départemental pourrait répondre à ce besoin, tout en étant particulièrement pertinente pour la compréhension fine du fonctionnement des dispositifs locaux de protection de l'enfance. Une vue d'ensemble, complète, des données des comités départementaux, apporter une vision plus précise sur les disparités- notamment de prise en charge -, qui demeurent importantes, contribuerait à l'harmonisation de ces politiques publiques décentralisées sur le territoire national, tout en diffusant de fait les bonnes pratiques. Notre amendement a donc pour objet de compléter les missions des comités départementaux

il n'a pas vocation à rédiger des rapports ou à faire des évaluations. C'est le travail de l'ODPE, qui est très utile et complémentaire. Le comité pourra d'ailleurs s'appuyer sur ces travaux d'expertise. Je rappelle à l'attention

Le comité chargé de coordonner les politiques et mettre en oeuvre des actions communes, notamment en matière de prévention, pourra déjà formaliser ces actions dans un tel projet, sans qu'il soit nécessaire de l'inscrire dans la loi. Il conviendrait en outre

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement a pour objet d'actualiser la dénomination des associations qui interviennent, depuis des années, en faveur des mineurs et jeunes confiés ou accueillis à l'aide sociale à l'enfance. En ce sens, il tend à modifier l'article L. 224-11 du code de l'action sociale et des familles, en favorisant de plus la pluralité des associations au sein d'un même département. En effet, nous nous trouvons actuellement dans une situation un peu absurde : certains départements comptent plusieurs associations, quand le droit

Nous proposons donc de remédier à cette absence de reconnaissance de la pluralité et de la diversité des associations, en espérant favoriser, d'ailleurs, l'émergence de nouvelles structures.

notamment grâce à sa regrettée vice-présidente Emmanuelle Ajon, s'est doté d'un conseil des jeunes de la protection de l'enfance, afin d'évaluer et d'améliorer régulièrement les dispositifs en cours dans le secteur. Celui-ci rencontre un véritable succès, et les nombreuses observations réalisées lors de la première mandature démontrent l'utilité de ces structures. Elles donnent un espace aux jeunes pour échanger, pour s'exprimer, pour agir, mais elles permettent aussi aux départements de se nourrir des retours des usagers que sont les enfants placés.

Avec un objectif similaire- vous en avez parlé, monsieur le secrétaire d'État -, le Haut Conseil aux enfants placés de l'Allier réunit régulièrement des jeunes placés ou anciennement placés pour évaluer et améliorer sa politique en s'appuyant sur la parole des premiers concernés. Ces initiatives et expérimentations, qui se sont montrées concluantes, doivent être encouragées pour être généralisées. Leur contribution à la conception et à la mise en oeuvre d'une politique publique pertinente et démocratique est essentielle.

entre les professionnels, ce qui me semble intéressant et important. Par ailleurs, ils ont dénoncé une forme de préjugés face aux enfants de l'ASE. On le voit, il s'agit d'une parole précieuse. Il serait donc bon de se servir de cette expérience pour la généraliser à l'ensemble des départements.

Plutôt que de créer une structure supplémentaire à côté de celles qui existent déjà, il me semble préférable d'associer, en lien avec les professionnels, les enfants et les associations d'anciens enfants protégés dans les structures de gouvernance actuelles : le nouveau GIP le prévoit et la gouvernance territoriale que nous proposons pourra également le faire.

l'avis du Gouvernement ? Depuis ma nomination, j'ai à coeur que soit mieux prise en compte la parole des enfants, pas uniquement celle des anciens enfants protégés, mais aussi celle des enfants qui sont actuellement confiés. C'est d'ailleurs

mais faisons confiance aux départements pour s'en emparer. S'il y a une valeur ajoutée, ils s'en empareront

d'une proposition de loi déposée par notre ancienne collègue Josiane Costes, vise à mieux protéger les adolescents arrivés sur notre sol au terme d'un parcours dangereux, qui se trouvent fragilisés par cette expérience et par l'absence de protection et de prise en charge par un adulte digne de confiance. Il s'agit de faciliter cette prise en charge par les services de l'enfance en instaurant une présomption d'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pour leurs parents résidant à l'étranger. Quel est l'avis de la commission ? Cet

et ne spécifie pas dans son dispositif qu'il ne s'appliquerait qu'aux MNA. L'adoption de cet amendement créerait donc une présomption de l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pour tous les parents se trouvant à l'étranger et ayant un enfant en France.

Il s'agit de garantir une plus grande équité entre les départements dans l'accueil des mineurs non accompagnés. Tenir compte des mineurs non accompagnés jusqu'à l'âge de 21 ans

Cet amendement tend à insérer une section spécifique consacrée aux conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.

constitue à bien des égards une réelle avancée dans la protection des MNA, puisqu'il a pour objet d'interdire les réévaluations très courantes des jeunes reconnus mineurs et isolés par un département. en effet que l'orientation du mineur, selon la clef de répartition nationale, repose toujours sur une décision judiciaire- parquet ou juge des enfants -, en application des alinéas 3 et 4 de l'article 375-5 du code civil. Ainsi, lorsque le département

que ces défauts d'exécution soient constatés et sanctionnés par les tribunaux administratifs. Encore faut-il que le mineur soit accompagné par des associations ou des avocats. Un département a cependant toujours les moyens de contourner les dispositions de cet article en faisant défaut de l'exécution de la décision du juge. C'est pourquoi il est nécessaire de renforcer les mesures mises en place par l'article. Est prévue à cette fin la possibilité pour le juge des enfants d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, mais cette possibilité de fait est rarement mobilisée en matière d'assistance éducative- c'est paradoxal. Cela constitue pourtant un moyen supplémentaire pour le juge qui constaterait des défauts d'exécution récurrents ou des délais excessifs, voire dilatoires, pour s'assurer de la bonne exécution de cette décision.

identique a donc pour objet de protéger réellement les mineurs non accompagnés contre les réévaluations en rappelant la possibilité d'ordonner des astreintes pour assurer l'exécution effective des décisions du juge à l'origine de l'orientation. La loi prévoit la possibilité pour le juge des enfants d'ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision, mais cette possibilité est rarement utilisée en matière d'assistance éducative. Cela constitue pourtant un moyen supplémentaire pour le juge qui constaterait des défauts d'exécution récurrents ou des délais excessifs de s'assurer de la bonne exécution de ces décisions. cette possibilité dans le cas des décisions d'orientation prises par les juges des enfants. Quel et 375 ont pour objet de rappeler que le juge des enfants peut prononcer une astreinte à l'encontre du département qui ne respecte pas sa décision concernant la reconnaissance d'un jeune comme mineur non accompagné. Si l'on peut regretter le manque d'application par certains départements des mesures ordonnées par le juge s'agissant des MNA, la loi permet déjà à celui-ci de prononcer des astreintes. En outre, l'article 14 interdit expressément aux départements de procéder à des réévaluations de la minorité.

Cet amendement vise donc à supprimer la compétence du parquet pour se prononcer sur l'orientation vers un département du jeune évalué comme MNA par un président de conseil départemental. Seuls les juges des enfants seraient alors compétents.

l'évaluation de la minorité (AEM) soit efficient, par l'instauration de sanctions financières. En effet, si un département n'organise pas la présentation des MNA et ne transmet pas tous les mois les décisions individuelles prises à l'issue des évaluations, la contribution forfaitaire de l'État pour la phase d'évaluation ne lui sera pas versée. Pour rappel, pour 100 MNA, la contribution forfaitaire s'élève à 50 000 euros.

L'article 15, de plus, ne relève pas d'une question de protection de l'enfance, mais davantage d'un enjeu de régulation des flux migratoires. Il met à mal la règle de présomption de minorité en nous faisant passer d'une évaluation « en cas de doute » à une évaluation généralisée, sauf en cas de minorité manifeste.

et ses droits à la protection priment. Cet article a été rédigé sans qu'aucune évaluation soit faite de l'usage du fichier AEM par les départements y recourant déjà de manière volontaire. Il a comme principale justification le nomadisme des mineurs isolés, petit frère- ou petite soeur -de la théorie de l'appel d'air. Or ces concepts ne sont ni validés ni étayés par aucune analyse sérieuse, ni ni quantitative ni qualitative. À défaut d'une réalité signifiante, ils relèvent d'une approche essentiellement idéologique. Ce qui est réel aujourd'hui, c'est que plus des deux tiers des enfants qui font un recours auprès d'un juge des enfants sont reconnus mineurs. Cette

législatifs, mais de protéger les enfants en danger, y compris en respectant la présomption de minorité. Toute autre politique serait contraire aux recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations unies. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article 15.

par l'article 39 de ce projet de loi, le recours à l'AEM. Cette disposition est ici reprise dans un projet de loi visant à protéger les enfants. Il n'existe pas de statut juridique propre aux mineurs isolés étrangers. Ces derniers se trouvent donc à un croisement relevant à la fois du droit des étrangers et des dispositions sur l'enfance en danger. Or le dispositif français de protection de l'enfance ne pose aucune condition de nationalité. C'est le statut d'enfant qui devrait prévaloir pour ces personnes, et non le statut d'étranger, conformément aux engagements de la France au titre de la Convention internationale des

est l'avis de la commission ? Je ne vais pas vous rappeler ce que l'article 15 prévoit de rendre obligatoire. Afin de rendre effectives les obligations, cet article prévoit également de conditionner à leur respect le versement de la contribution forfaitaire de l'État aux départements.

Un tel fichier national permet d'éviter le phénomène de nomadisme de la part de majeurs qui tentent leur chance dans différents départements et engorgent les dispositifs d'accueil. La généralisation de ce fichier au niveau national apparaît comme nécessaire pour accroître son efficacité et améliorer la qualité des évaluations dans tous les départements.

Le département a reçu compétence pour mener à bien l'évaluation. Et le mineur qui est évalué majeur

des enfants. Cet amendement vise à replacer le juge des enfants comme acteur central de la procédure d'évaluation chargée de déterminer, avec l'appui des départements et des services de l'état le cas échéant, en même temps que l'existence d'un danger ou d'un risque de danger, si la personne est mineure ou non - conformément aux articles 375 et suivants du code civil. Cet amendement prévoit l'ordonnance de mesures provisoires par le juge des enfants lorsque celui-ci est saisi sans délai par le service auprès de qui le mineur se déclarant privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est présenté, et le maintien de l'accueil provisoire d'urgence tant que la décision du juge n'intervient pas. La compétence du parquet pour prendre des mesures provisoires ne peut en principe être exercée qu'en cas d'urgence grave, en dehors du temps de présence au tribunal du juge des enfants. Concernant les MNA, elle est utilisée systématiquement, alors qu'en réalité les conditions de son exercice ne sont pas remplies. Dans la grande majorité des cas, le département et le parquet sont les seuls à statuer sur la minorité et l'isolement des mineurs isolés qui ne sont pas encore en capacité d'exercer un recours. Cet amendement rétablit donc le rôle central du juge des enfants. Ce dernier est souverain dans son appréciation de la majorité ou de la minorité. Il peut ordonner les examens selon la procédure définie dans le code civil. Cela permet de mettre un terme aux ruptures de protection et à la violation des droits fondamentaux des mineurs dont les départements refusent l'admission à l'aide sociale qui sont souvent reconnus, sur décision du juge des enfants après plusieurs mois passés sans protection. Il s'agit aussi de se mettre en conformité avec le droit international et la jurisprudence. Cet amendement a pour objet, à cet effet, de réaffirmer qu'un jeune se présentant comme mineur doit être considéré comme tel jusqu'à ce qu'une décision de justice

: La parole est à M. Roger Karoutchi. Lorsque l'intéressé n'est pas en possession d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité du pays d'origine, il paraît opportun d'exiger que les documents d'état civil produits soient légalisés, conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 2019. L'évaluation par les investigations prévues par l'article 15 du projet de loi ne revêtirait qu'un caractère subsidiaire, dans les cas où le mineur a établi qu'il est dans l'incapacité de présenter des documents authentifiés, qu'il a effectué des démarches en ce sens qui n'ont pas encore abouti, ou que sa minorité est manifeste. Cet amendement supprime le dixième alinéa de l'article 15 du projet de loi, qui ne paraît pas nécessaire puisque le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont déjà consacré le principe selon lequel la majorité d'une personne ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes ou de son seul enregistrement dans le fichier AEM. Enfin, cet amendement supprime le renvoi à un décret en Conseil d'État de la fixation de la durée de l'accueil provisoire d'urgence. Cette durée varie considérablement d'un département à l'autre. Il ne paraît donc pas opportun de réglementer de manière uniforme la durée de l'accueil provisoire d'urgence, cette durée n'ayant pas, en tout état de cause, de caractère obligatoire.

nous a été, lui aussi, inspiré par Unicef France. Il a pour objet de rétablir le renvoi essentiel aux dispositions relatives à l'accueil provisoire d'urgence, tel que le prévoit aujourd'hui la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles. En effet, l'article 15, dans sa réaction actuelle, supprime le renvoi, pourtant essentiel, à l'article L. 223-2 de ce code. L'inscription de l'accueil provisoire d'urgence dans la partie législative de ce code est primordiale. En effet, les MNA sont d'abord des mineurs privés de leurs représentants légaux, et l'administration ne peut maintenir sous sa protection des enfants sans l'accord de leurs représentants légaux de manière indéfinie. Il est primordial que leur situation juridique soit sécurisée par l'intervention de l'autorité judiciaire, même lorsque l'évaluation se poursuit. Alors que de nombreux départements ne mettent pas en place cet accueil, ou le diffèrent malgré un cadre légal contraignant - ils sont d'ailleurs condamnés pour cette raison -, il est à craindre que cette suppression du renvoi à l'article L. 223-2 renforce encore ces carences. C'est également ce qu'observe la Défenseure des droits, qui indique que « ce nouvel article prévu par le projet de loi viendrait conforter de façon très inopportune les pratiques juridiquement contestables des départements qui ne respectaient pas l'article L. 223-2 du code de Cet amendement tend également à rétablir les dispositions qui prévoient le maintien de l'accueil provisoire d'urgence tant que la décision de placement provisoire de l'autorité judiciaire n'intervient pas. Finalement, cet amendement relève du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant,

MNA, de décembre 2019, suggère qu'il est pertinent de permettre à la personne de bénéficier d'un temps de répit lors de son accueil et préalablement - j'y insiste -au début de la procédure d'évaluation de sa situation. d'évaluation de sa situation. Ce temps peut contribuer à éviter que l'évaluation repose sur des éléments recueillis sur des mineurs en souffrance, épuisés, parfois en errance psychique, et donc incapables d'apporter des réponses détaillées et cohérentes, notamment concernant leur parcours de vie.

pour établir l'identité d'une personne. De même, l'article 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) consacre le droit à l'identité du mineur, en prévoyant la reconnaissance des documents d'état civil présentés.

La circulaire du 1 avril 2003 précise pourtant que la force probante d'un acte de l'état civil étranger doit être retenue dès lors que sa régularité formelle n'est pas contestée. Mais cette disposition n'est pas respectée.

Il est également courant que les autorités administratives ou judiciaires disqualifient les documents présentés par les jeunes demandeurs au motif qu'ils ne comportent pas de photographie, et qu'il est donc impossible de confirmer l'appartenance de l'acte au jeune. Enfin, il est rare qu'au stade de l'évaluation, les services qui en sont chargés accompagnent les intéressés dans la reconstitution de leur état civil lorsque celui-ci est absent, alors même que cette reconstitution est explicitement prévue à l'article 8 de la CIDE. Cet amendement rappelle donc ces principes et définit les conditions dans lesquelles la présomption d'authenticité des documents d'état civil peut être renversée, ainsi que la façon dont le département peut assister le mineur dans la reconstitution de son état civil. L'amendement Mme Raymonde Poncet Monge. Outre les dispositions relatives à d'usage du fichier AEM, l'article 15 prévoit que le conseil départemental peut demander à l'autorité judiciaire de recourir aux tests osseux dans le cadre de l'évaluation de minorité. cet usage des tests osseux est à proscrire. En effet, les planches de référence qui servent à analyser par tranche de six mois l'évolution des os du poignet ont été réalisées en 1930. À l'époque, leur objectif n'était pas de déterminer l'âge des mineurs, mais d'analyser la croissance des enfants.

de solliciter un médecin pour pratiquer et interpréter un test qui n'est pas validé scientifiquement et qui, en outre, n'est pas mis en oeuvre dans l'intérêt thérapeutique de la personne (CNCDH), la Défenseure des droits et toutes les autorités consultatives plaident pour que l'on interdise, comme au Royaume-Uni, cette gabegie d'examens. On parle quelquefois d'examens inutiles. En voici un ! L'évaluation de la minorité doit être le fruit d'entretiens

Cet amendement a pour objet de préciser que la présentation des mineurs non accompagnés en préfecture et le recours au fichier AEM n'ont lieu qu'en l'absence de documents d'état civil valables. Il permet de réaffirmer le principe de la présomption d'authenticité des documents d'état civil, posé par l'article 47 du code civil. Il s'agit bien entendu d'un amendement de repli, puisque nous sommes favorables à la suppression de l'article 15

rendre obligatoire la présentation auprès des services préfectoraux de la personne se présentant comme mineur non accompagné, afin que ceux-ci apportent une aide à l'identification et à l'évaluation de la minorité par la consultation du fichier AEM. Le président du conseil départemental n'est toutefois pas tenu à cette présentation lorsque la minorité de la personne est manifeste. Cette rédaction nous semble imprécise. Aussi, nous proposons que la présentation des MNA en préfecture et le recours aux fichiers AEM aient lieu en cas de doute sur la minorité, et non plus « sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste ». Cette rédaction fait par ailleurs écho aux termes employés dans l'article 388 du code civil.

L'amendement n° 21 rectifié vise à centrer l'évaluation de la minorité sur la possession par l'intéressé de documents d'état civil légalisés, et à rendre subsidiaires les autres investigations, notamment sociales et psychologiques. Les MNA provenant en grande majorité de pays où l'état civil n'est pas tenu correctement, une telle mesure nécessiterait que tous les jeunes ou presque entament des démarches auprès des autorités consulaires, sans certitude de résultat, ce qui allongerait considérablement et inutilement les délais d'évaluation. En outre, les entretiens réalisés avec le jeune gardent toute leur pertinence pour évaluer l'isolement de ce dernier. En conséquence, l'avis est défavorable.

Ils prévoient que le président du conseil départemental se doit, dès le stade de l'évaluation, d'assister les jeunes dans leurs démarches auprès des autorités consulaires. Ils ne semblent toutefois pas applicables en pratique et risqueraient d'allonger considérablement les délais d'évaluation. L'avis est donc défavorable. Les amendements n 373 et 292 fixent à cinq jours la durée de l'accueil provisoire d'urgence du jeune à l'issue de laquelle le président du conseil départemental doit saisir l'autorité judiciaire,

de retrouver leurs esprits avant le début des entretiens. S'il est prévu par le guide de recommandation des bonnes pratiques en matière d'évaluation, il est rarement appliqué par les départements. Il serait donc opportun de l'inscrire dans la loi. Avis favorable, Les amendements n 367 rectifié et 288 proposent de supprimer le fichier d'aide à l'évaluation de la minorité, tandis que l'amendement n° 42 rectifié vise à supprimer le recours obligatoire à ce fichier. Pour les mêmes raisons que celles que j'ai développées sur les amendements de suppression de l'article 15 tout à l'heure, l'avis est défavorable.

entend conditionner le recours au fichier AEM à l'existence d'un doute sur la minorité. Cette condition est équivalente à la condition actuelle, qui prévoit que la consultation a lieu

vise à supprimer la possibilité de recourir aux tests osseux. Il s'agit d'une méthode facultative parmi les nombreuses qui concourent à l'évaluation de la minorité. Elle ne peut être réalisée qu'en saisissant l'autorité judiciaire et dans le respect de règles strictes rappelées par le Conseil constitutionnel.

de séjour. L'amendement ouvre toutefois cette possibilité au stade de l'évaluation, c'est-à-dire pour des personnes qui ne sont pas encore reconnues mineures et dont certaines, une fois majeures, seront soumises à une obligation de quitter le territoire français.

tous les actes de l'autorité parentale pendant la phase de l'évaluation de minorité- autorisation de soin, autorisation de pratiquer un sport, autorisation de passer les tests nécessaires à la scolarisation, autorisation de droit de visite et d'hébergement chez un tiers, etc. Quel

En 2016, le Défenseur des droits avait ainsi affirmé que la scolarisation des jeunes migrants devait être une priorité absolue. C'est pour atteindre cet objectif que notre amendement prévoit d'organiser la scolarisation des mineurs non accompagnés, avec, dès leur accueil provisoire, l'évaluation de leur niveau scolaire et leur affectation dans un établissement.

a ainsi montré que l'os sésamoïde du pouce pouvait apparaître entre 10 et 15 ans chez les garçons et entre 8 et 15 ans chez les filles. Nous utilisons donc un test dont la marge d'erreur,

. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de recourir aux tests osseux pour établir la minorité des mineurs non accompagnés. Rappelons tout d'abord- tout le monde le sait ici -que le référentiel relatif aux tests osseux date de 1930. Il semble donc légèrement dépassé Qu'elle soit prise isolément ou combinée, aucune méthode médicale de détermination de l'âge osseux n'apporte, à l'heure actuelle, des informations scientifiques suffisamment fiables et précises pour déterminer l'âge des mineurs évalués.

pour procéder à l'évaluation de la minorité lorsque l'intéressé se déclare mineur et privé temporairement, ou définitivement, de la protection de sa famille. Par ailleurs, la présomption de minorité dont bénéficie l'intéressé jusqu'à ce que l'évaluation de son âge ait été réalisée est consacrée par cette proposition.

comme mineure soit considérée comme telle jusqu'à ce qu'une décision de justice ayant autorité de la chose jugée, donc une décision du juge des enfants ou de la cour d'appel, soit rendue.

Comme l'indique la Cimade dans son avis sur le projet de loi que nous discutons aujourd'hui, le recours au fichier d'appui à l'évaluation de la minorité « met en avant un contrôle et une gestion des flux migratoires inconciliable avec la protection de l'enfance. Cette disposition renverse d'ailleurs la présomption de minorité et le bénéfice du doute. De plus, l'enregistrement des données personnelles des enfants à d'autres fins que celles liées à leur protection est manifestement contraire aux recommandations du comité des droits de l'enfant ». La présomption de minorité ne peut être écartée lorsque celle-ci n'est pas manifeste. Il s'agit d'un principe absolu auquel nous voulons aujourd'hui donner, par cet

18 rectifié est satisfait par l'article 15, qui prévoit que le président du conseil départemental procède à l'évaluation. Sur le second point, il n'apparaît pas nécessaire d'inscrire une présomption de minorité dans la loi, alors que tout jeune se déclarant MNA arrivant en France bénéficie d'un accueil provisoire d'urgence, le temps d'être évalué. De plus, si, à l'issue de l'évaluation, il subsiste un doute sur son âge, celui-ci profite à la personne. Une présomption de minorité n'apporterait donc aucune garantie supplémentaire. La commission demande donc le retrait de cet amendement

afin de prévoir, dans les cas où il existe un doute sur la minorité de la personne pour laquelle il est envisagé de prendre des mesures d'assistance éducative, que l'autorité judiciaire saisisse le président du conseil départemental afin qu'il procède à l'évaluation de la minorité dans les conditions prévues par la loi. Les exigences de sécurité juridique et d'efficacité imposent que les différentes autorités chargées de déterminer si une personne se déclarant mineure doit bénéficier du dispositif de protection de l'enfance ne prennent pas des décisions contradictoires sur la question de la minorité de la personne. En outre, eu égard aux qualifications exigées par les dispositions réglementaires applicables aux travailleurs sociaux chargés de procéder à l'évaluation de la minorité mise à la charge des départements, il apparaît opportun que le juge des enfants saisi en application de l'article 375 du code civil puisse, pour prendre une décision éclairée, bénéficier de l'expertise des services du département spécialement formés à cet effet.

Fodé Traoréiné, arrivé en France après ses 16 ans, s'est vu remettre une OQTF à sa majorité, alors qu'il était en passe de valider son certificat Son patron est allé jusqu'à faire une grève de la faim pour que son apprenti soit régularisé et une pétition en ce sens a réuni plus de 240 000 signatures. En 2015, Armando Curri, titulaire d'un CAP de menuiserie désigné meilleur apprenti de France ici même au Sénat, avait fait l'objet d'une OQTF quelques mois auparavant, au point que la cérémonie a failli ne pas avoir lieu. Ces histoires absurdes ne sont pas des cas isolés ; elles se répètent dramatiquement, régulièrement. année 2021, la Cimade accompagnait à elle seule près de 200 anciens MNA visés par des OQTF. Comment comprendre qu'un mineur ayant fait l'objet de mesures de protection, d'accompagnement, de soutien par les services de l'ASE puisse, du jour au lendemain, se retrouver à la porte d'un système qui a pourtant, et à raison, tout entrepris pour garantir son intégration ? Ce gâchis doit cesser. Les MNA qui ont été pris en charge par l'ASE doivent, de droit, recevoir à leur majorité Il s'agit de faire oeuvre de cohérence administrative et de respecter le travail de l'aide sociale à l'enfance, le travail des travailleurs sociaux, l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de ces jeunes à poursuivre leur intégration dans notre pays. L'amendement

vise à sécuriser les parcours des jeunes majeurs ex-MNA et de permettre leur admission au séjour mention « vie privée et familiale », quel que soit l'âge auquel ils ont été confiés à l'ASE. En effet, la carte de séjour « vie privée et familiale » est une condition essentielle de l'insertion sociale et professionnelle. Contrairement à la carte « travailleur temporaire » actuellement délivrée aux jeunes pris en charge après 16 ans, cette carte de séjour marque le caractère pérenne de la présence du jeune sur le territoire ; elle permet un accès au marché de l'emploi

ASE est la date de la mise à l'abri- cette modification permet de ne pas pénaliser le jeune pour les délais inhérents à l'évaluation de minorité et à l'obtention de en supprimant la possibilité d'accorder une carte « travailleur temporaire », qui ne donne pas accès au contrat d'intégration républicaine et qui marque le caractère temporaire de l'admission au séjour des jeunes majeurs ex-MNA, en l'espèce le temps du contrat de travail. Quel

Comme l'amendement n° 222 rectifié, il permet aussi aux MNA d'obtenir de plein droit une carte de séjour « vie privée et familiale », quel que soit l'âge auquel ils ont été pris en charge par l'ASE, alors que cette possibilité est ouverte aux seuls MNA confiés à l'ASE avant 16 ans.

le taux d'approbation des demandes de titre de séjour est très élevé : plus de 90 %. Je vous propose donc de rester sur cette approche et de ne pas modifier les conditions d'obtention d'une carte de séjour, compte tenu des

L'obtention d'une carte de séjour « salarié » pour les anciens MNA arrivés en France après 16 ans relève d'une procédure d'admission exceptionnelle au séjour, c'est-à-dire dérogatoire aux conditions d'obtention dont bénéficient les autres étrangers. Le pouvoir d'appréciation de l'administration est plus grand. La suppression de ce caractère exceptionnel n'aurait pas d'influence sur les conditions d'obtention ni sur les marges de manoeuvre de l'administration. Elle n'apparaît donc pas nécessaire. ailleurs, la carte portant la mention « travailleur temporaire » est délivrée aux étrangers détenant un CDD. Cette règle s'applique à tous les étrangers, et instituer une distinction pour les anciens MNA ne semble pas être justifié. La commission émet donc un avis défavorable

en vertu de l'article 388-1-1 du code civil, « l'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes Or les mineurs non accompagnés sont, par définition, sans représentant légal sur le territoire, tant qu'ils n'ont pas été reconnus mineurs et qu'une décision judiciaire n'a pas déféré leur tutelle au président du conseil départemental. Il paraît primordial qu'ils bénéficient d'une représentation légale dès leur entrée sur le territoire, afin que puissent être effectués tous les actes de la vie civile les concernant, qu'ils puissent être accompagnés dans toute procédure, y compris la procédure d'évaluation de leur minorité, et de pallier les difficultés d'accès à la justice qu'ils peuvent rencontrer. C'est pourquoi cet amendement proposer que le Gouvernement remette au Parlement, suivant la formule consacrée, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la désignation systématique d'un administrateur pour tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille.

l'attention sur la situation de crise et d'urgence que connaît l'aide sociale à l'enfance, notamment au travers du métier d'assistant familial, et sur le devenir

Aujourd'hui, si un éducateur de l'ASE souhaite devenir famille d'accueil, il lui faut soit se mettre en disponibilité, soit démissionner, car il ne peut pas cumuler le statut de fonctionnaire et le statut de contractuel de la fonction publique. Or il pourrait être intéressant que des professionnels

des enfants et des professionnels -, au délai de trois mois pour le retour sur les informations préoccupantes ou encore à la réécriture de l'article 3 D afin de protéger davantage les jeunes majeurs.

Ce texte constitue une avancée très importante dans la prise en charge de l'enfance par l'ASE. Je voudrais féliciter le rapporteur, Bernard Bonne, qui s'est beaucoup impliqué

ce qui nuit gravement à la prise en charge des enfants de l'ASE. Nous regrettons le rejet de l'amendement présenté par Colette Mélot qui visait à inscrire la prévention et la lutte contre la prostitution des mineurs dans une stratégie de prévention. Les faits de prostitution sont extrêmement graves et nous devons identifier et réprimer avec une grande fermeté les auteurs de ces actes. Dans l'ensemble, le projet de loi contient des avancées importantes : l'interdiction de placement en hôtel, le droit de retour des enfants à l'ASE jusqu'à 21 ans, le renforcement du contrôle des antécédents judiciaires des personnels, le parrainage et le mentorat, et surtout la sécurisation du métier d'assistant familial avec l'augmentation des salaires, la formation et la participation à l'élaboration du projet des enfants. Par conséquent, notre groupe votera ce projet de loi.